régions. Pour l'année 2020, le Groupement des autorités responsables de transport, qui réunit plus de 200 autorités organisatrices de la mobilité, estime que celles-ci feront face à une baisse de 10 % des recettes liées au versement mobilité,

cadre du PLFR 4, le Gouvernement a prévu un mécanisme d'avances remboursables pour compenser les pertes commerciales, à hauteur de 750 millions d'euros : un geste fort pour les AOM, qui mérite d'être salué. Cependant, rien n'est prévu pour compenser les pertes liées à la baisse du versement mobilité, qui peut représenter, parfois, près des trois quarts des recettes des AOM-

présent amendement, nous proposons que cette double couverture des pertes- versement mobilité et recettes commerciales -soit étendue à l'ensemble du pays. Il s'agirait de créer un fonds à hauteur de 750 millions le même montant que les avances remboursables précédemment accordées -afin de soulager la situation financière inquiétante des AOM. Cela répondrait à un impératif de justice et d'égalité entre les territoires. Quel

Cette discussion commune est liée au fait que ces amendements, traitant de thématiques variées, prélèvent des crédits sur l'action n° 01, Financement des entreprises, du programme 363, « Compétitivité ». Le montant cumulé de ces prélèvements serait très supérieur aux crédits inscrits à cette action.

La crise sanitaire entraîne une crise sociale dramatique, avec une explosion des inégalités et une fracturation de la société. Il y a urgence à aider les plus démunis, en augmentant significativement

les organisations syndicales, mais également Esther Duflo, prix Nobel d'économie en 2019. Toutes et tous exigent une revalorisation du revenu de solidarité active, ainsi que son ouverture aux jeunes dès 18 ans. En 2020, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de près de 10 %.

comme le rapporte le Secours catholique, des centaines de milliers de ménages se sont retournés vers les associations caritatives et les collectivités territoriales pour solliciter une aide alimentaire ou financière. Affectés par une brutale perte de revenus ou une hausse de leurs dépenses- parfois les deux les deux -, ils viennent de basculer dans une situation d'extrême urgence. Parmi ces personnes et ces familles, on trouve de nombreux allocataires de minima sociaux. Pour pallier l'insuffisance des prestations sociales pendant le confinement, le Gouvernement avait opté pour une prime unique de 150 euros accordée aux bénéficiaires de minima sociaux. Les associations considèrent cette mesure comme dérisoire et regrettent, face à l'ampleur des difficultés structurelles rencontrées par les ménages, l'absence de revalorisation de ces minima. En effet, contrairement aux dires d'Emmanuel Macron, l'augmentation des minima sociaux permettrait aux bénéficiaires de se consacrer davantage à la recherche d'un emploi. C'est pourquoi nous proposons, avec cet amendement d'appel, de financer une revalorisation des minima sociaux à hauteur de 500 millions d'euros. L'amendement

Ils ont vécu avec d'énormes difficultés la rentrée de septembre, puis le reconfinement, et on leur annonce, maintenant, que les universités ne seront pas rouvertes avant février, voire plus tard. Il faut absolument, monsieur le ministre, que vous entendiez la grande détresse des étudiants. Il faut se préoccuper de cette jeunesse, dont la situation est catastrophique et qui a le sentiment de constituer la génération sacrifiée de la pandémie.

dans le monde universitaire. Je ne peux pas laisser dire que rien n'a été fait, loin s'en faut ! L'avis est donc défavorable sur ces deux amendements.

de la recherche. Or, dans aucun de ces textes, à aucun moment, il n'a été question de la vie étudiante, hormis les quelques mesures que vous avez indiquées, qui vont dans le bon sens, mais concernent les seuls boursiers.

je connais de notre économie nationale, et en l'état actuel des choses, une grande part de l'activité du pays est liée au niveau de consommation intérieure. Donc,

Si nous ne donnons pas du pouvoir d'achat aux catégories les plus populaires, notamment à la jeunesse et aux étudiants- qui ne vont pas s'empresser d'aller remplir leur livret d'épargne -, nous n'aurons pas le niveau de consommation intérieure nécessaire et souhaitable.

vise donc à soutenir l'investissement des collectivités locales, sachant que, en termes d'investissement local, près de 60 % de la commande publique relève des commandes de ces collectivités. Les régions bénéficient déjà de 600 millions d'euros

Merci,

de loi de finances, des mesures fortes de soutien financier aux collectivités ont été adoptées, permettant, selon moi, d'accroître leurs capacités d'autofinancement et, donc, d'investissement. Pour ces raisons, je demande le retrait

Au total, de janvier à août 2020, leur chiffre d'affaires a chuté de 37 %. En novembre, leur activité a de nouveau diminué de 60 %, selon l'Insee. Les aides d'urgence mises en place par l'État permettent, certes, le paiement des charges de personnel et offrent une forme de répit de courte durée pour la trésorerie de ces entreprises, mais elles ne couvrent pas l'ensemble des dépenses : stocks, loyers, salaires de l'employeur, autres charges fixes, etc. creuseront leur endettement et détérioreront leur solvabilité, déjà fragile. Au-delà des aides d'urgence, aucune mesure du plan de relance du Gouvernement n'est spécifiquement dédiée à ce secteur, alors même que sa situation dramatique est régulièrement au centre du débat public depuis plus de huit mois. Le plan pour l'économie de proximité se concentre, par exemple, sur la rénovation de locaux vacants et le développement ou le financement de solutions numériques, certes utiles, mais qui ne peuvent suffire. Parallèlement, et de façon générale, le plan de relance du Gouvernement manque de mesures spécifiquement dédiées à la demande, notamment à celle des plus modestes, qui ont pourtant une propension marginale à consommer élevée. Or, une fois la réouverture des restaurants autorisée, c'est bien à un risque d'insuffisance de la demande que ces derniers feront face. Durant l'été postérieur au premier confinement, par exemple, le marché de la restauration n'avait atteint que 70 % du chiffre d'affaires enregistré au cours de l'été 2019. Cet amendement vise donc à créer un fonds doté de 400 millions d'euros, permettant la prise en charge par l'État, pour une durée d'un mois, de chèques-restaurants à destination des ménages les plus modestes, dans le but de soutenir leur consommation et de relancer le secteur de la restauration lors de sa réouverture. Ces chèques Ces chèques seraient distribués par les communes volontaires, par exemple, les centres communaux d'action sociale, qui ont une forte légitimité en la matière. Les restaurateurs se feraient rembourser auprès de ces organismes le montant des chèques dépensés dans leur établissement, la commune obtenant ensuite

le cadre de l'accord en commission mixte paritaire sur la loi de programmation de la recherche, notre brillant collègue Jean-François Rapin, rapporteur spécial des crédits de la mission

J'ai écouté religieusement la réponse du ministre des outre-mer hier : entre les paroles et les actes, franchement ... Quand ça arrange certains, les outre-mer, c'est la France

a sollicité Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques, qui elle-même m'a demandé d'organiser, en tant que rapporteure pour avis du budget de la politique de la ville, une audition des maires ayant signé une lettre au Président de la République, le 14 novembre

quartiers prioritaires de la politique de la ville sur leur territoire. Ce fonds devrait leur permettre de faire face à l'urgence sociale qui résulte de la crise, d'amorcer les projets de développement local

arriver à prouver qu'on met 1 % des dépenses publiques dans un plan pour tel ou tel territoire est un exercice technique qui n'est pas difficile : il suffit de prendre en compte telle baisse de TVA ou telle subvention, d'ordre général,

: voilà des années qu'on explique que la politique de la ville s'enlise dans cette bureaucratie, délégitimant l'intervention publique. Ils n'en peuvent plus ! Aujourd'hui, ils nous demandent

présente, où les maires ont du mal à la défendre. Les problèmes sociaux sont tellement importants qu'aujourd'hui ceux-ci craignent de ne plus y parvenir. C'est un appel de détresse. J'ai compris, monsieur le rapporteur, que vous ne pourrez pas tout financer.

affaire, il y aurait, d'un côté, les mauvais petits canards, les parlementaires qui tentent d'exprimer des priorités, de faire valoir des points de vue, et, de l'autre, l'ange blanc

est à M. Éric Bocquet. Le 12 novembre dernier, M. le ministre de l'éducation nationale déclarait, dans le cadre du point d'étape du reconfinement : « Nous allons amener plus de jeunes du service civique, des assistants pédagogiques et des professeurs remplaçants.

en 2021. Cette somme doit financer 8 000 recrutements en 2020, ainsi que le recrutement de 4 000 AESH supplémentaires pour l'année scolaire 2021-2022 pour l'année scolaire 2021-2022 afin de répondre aux prescriptions des MDPH en matière d'aide à la personne. D'autre part, le PLF pour 2021 intègre une hausse de 31 millions d'euros des crédits prévus au titre de la rémunération des assistants d'éducation.

à Mme Laurence Cohen. Le présent amendement vise à proposer l'instauration d'un dispositif d'aide à l'installation de centres de santé. La crise sanitaire actuelle de la covid-19 est présentée par les scientifiques comme la première d'une série de futures pandémies, en lien avec le réchauffement climatique, notamment, selon une étude publiée par l'Unesco en octobre dernier. Dès lors, nous devons pallier le problème des déserts médicaux qui s'étendent dans les zones rurales comme dans les zones urbanisées. Notre groupe propose entre autres solutions l'installation sur tout le territoire de centres de santé publics. Ces centres offrent une structure d'exercice collectif coordonné salarié pour les jeunes médecins pour qui l'activité libérale n'est plus attractive,

En 2019, on évaluait à seulement 12 % le nombre de jeunes futurs médecins se lançant dans l'aventure libérale, tandis que 47 % d'entre eux choisissaient l'exercice salarié. Les centres de santé leur apportent une réponse pour la pratique d'une médecine globale et sociale centrée sur le patient, en lien avec tous les acteurs de leur territoire.

notre pays d'un tel outil, nous pourrions nous donner les moyens de produire sur notre territoire les masques de protection qui ont manqué hier, les tests de dépistage indispensables aujourd'hui et assurer, demain, la production et la distribution d'un vaccin, par exemple contre la covid-19, en ayant recours à la licence d'office. Cette discussion aura lieu le 9 décembre, et je ne doute pas qu'elle sera riche,

de retrouver une maîtrise publique de la production et de la distribution de médicaments ; ce pôle public est l'outil qui nous fait cruellement défaut Madame la sénatrice Cohen, 501 millions d'euros sont prévus pour sécuriser l'approvisionnement de la France en biens et produits médicaux jugés indispensables et concourant au maintien de sa souveraineté. C'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer

Ce second confinement est, pour nombre de ces entreprises, un coup fatal. Cet amendement d'appel vise à créer un fonds de sauvegarde qui s'appliquerait jusqu'au 30 juin 2021 afin de compenser leurs charges fixes, notamment les loyers, qui pèsent fortement sur elles. Ce mécanisme de Ce mécanisme de compensation des charges fixes serait indexé sur le niveau de reprise du chiffre d'affaires par rapport au niveau de l'année 2019, les éventuelles autres mesures d'aides touchées par l'entreprise seraient déduites du montant de cette compensation. Il permettrait d'assurer la simple survie de ces espaces de loisirs, tout en diminuant progressivement le soutien de l'État jusqu'au retour à un niveau d'activité égal à 80 % du chiffre d'affaires de 2019. Quel est l'avis de la commission ?

euros par mois, avec des loyers très importants, atteignant plus de 30 % du coût d'exploitation. Il est vrai que le Président de la République a pris une nouvelle série de mesures

Les PEC constituent depuis 2018 la nouvelle formule des contrats aidés ciblés sur le secteur non marchand. Ils apparaissent comme un outil efficace et rapidement mobilisable.

entretien et sa maintenance représentent un enjeu majeur en termes de sécurité routière, d'amélioration de la qualité de l'air et de pouvoir d'achat des automobilistes. En effet, une maintenance préventive des véhicules permet de limiter leur niveau d'émissions polluantes, de réduire les risques de panne et de réparations lourdes et de maintenir les véhicules dans des conditions optimales de fonctionnement

opérer un retrait de 110 millions d'euros sur le programme 363, « Compétitivité », avec 55 millions d'euros à l'action n° 02, Souveraineté technologique et résilience, et 55 millions d'euros à l'action n° 04, Mise à niveau numérique de l'État. Cette répartition permet de favoriser l'entretien et la réparation automobile dans une logique environnementale, car, au-delà de la seule pollution de l'air, les voitures qui ne sont pas entretenues souffrent de fuites

l'action économique de l'État.

En effet, la crise sanitaire et les quelque 85 % de projets désormais validés par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine font apparaître une importante demande d'amélioration et de complément des projets en cours. Le Président de la République l'a reconnu dans son discours aux Mureaux. Pour répondre à cette attente, 1 milliard d'euros d'investissements sont nécessaires. Afin de les amorcer et de solliciter les autres financeurs du programme, il convient que l'État assume sa quote-part, qui s'élève à 10 %, comme actuellement dans le nouveau programme national de renouvellement urbain. Quel

Personne n'est méprisé, personne n'est infantilisé, personne n'est soumis à je ne sais quel diktat ou oukase. Simplement, être responsable implique de tenir compte des conséquences de ses actes. Au fur et à mesure de ces votes,

de la gauche sénatoriale sont adoptés, cela démontre que cet avis sur les insuffisances du plan de relance est largement partagé.

à un équilibre. La grande priorité des maires, c'est d'avoir de l'argent pour les activités éducatives, l'éducation populaire et la présence associative, bref, de l'humain. La formation et les emplois aidés, c'est de l'humain

actuellement, le plan de relance, dans son volet biosécurité et bien-être animal en élevage, ne prévoit pas un soutien suffisant et ciblé à la transition des modes de production très intensifs- élevage en cage, sur caillebotis surdensité -vers des élevages respectueux des animaux, tels que les élevages au pâturage, le porc sur paille ou encore les poulets en plein air. Les investissements nécessaires à ces modes de production sont un vrai frein pour les agriculteurs qui souhaitent améliorer les conditions d'élevage. Par exemple, pour le porc sur paille, si, sur le terrain, de nombreux éleveurs souhaitent amorcer une transition et quitter le mode d'élevage sur caillebotis, les montants des investissements nécessaires sont bien souvent dissuasifs. Ces modes d'élevage respectueux du bien-être animal sont réclamés par nos concitoyens et sont également plus vertueux sur le plan environnemental.

commission ? La mission « Culture » intègre déjà cette problématique, puisqu'elle inclut la montée en charge du Fonpeps et la mise en oeuvre d'un plan dédié aux artistes-auteurs. Les entreprises culturelles ont par ailleurs accès à des dispositifs transversaux, à des degrés divers. Je demande donc le retrait

La collectivité calédonienne est un territoire particulièrement vulnérable face à la pandémie de covid. Des mesures strictes de fermeture des frontières et de suspension de la desserte aérienne sont prévues jusqu'en juillet prochain et une mesure de quatorzaine systématique s'applique pour tout nouvel arrivant sur son sol.

de l'AFD. La loi du 9 juillet 2020 relative à la sortie de l'état d'urgence a établi que la décision d'application de la quatorzaine relève de la compétence de l'État, et ce dans le respect de la répartition des compétences, telle qu'elle résulte de l'accord de Nouméa de 1998. L'État étant donc compétent en matière d'urgence sanitaire, le ministre des outre-mer s'est engagé, lors de sa venue, à ce que le Gouvernement prenne à sa charge les 75 millions d'euros de dépenses directement liées à la crise sanitaire, notamment pour le

Le soutien de l'État à la politique menée par la Nouvelle-Calédonie repose d'ores et déjà sur un prêt garanti par l'État, à hauteur de plus de 28 milliards de francs Pacifique, c'est-à-dire 230 millions d'euros.

pour présenter l'amendement n° II-263 rectifié . Le secteur du réemploi solidaire a été touché de plein fouet lors du premier confinement. Ses pertes nettes sont estimées à plus de 50 millions d'euros, malgré le chômage partiel et les aides du fonds de solidarité. Pour permettre à ces associations d'affronter la deuxième vague, le second confinement et les suites territoriales et nationales de la crise en 2021 et 2022, le renforcement du plan de relance à leur endroit devient plus que nécessaire, pour des raisons autant sociales qu'écologiques. Cet amendement vise donc à abonder le fonds Économie circulaire de l'Ademe de 75 millions d'euros sur deux ans, destinés exclusivement aux structures de l'économie sociale et solidaire, structures qui soutiennent l'insertion des plus précaires et la lutte contre le gaspillage, et réduisent les inégalités. La parole

visant à soutenir un secteur malmené par les deux confinements. Les organisations chiffrent à plus de 120 millions d'euros leurs pertes pour cette année. Le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le ministre, semble méconnaître l'importance de ce secteur pour l'emploi local, l'insertion et l'inclusion. Dans ma région des Pays de la Loire, sachez que l'économie sociale et solidaire représente près de 15 % de l'emploi : cela n'est pas un petit sujet économique. Ce secteur mérite d'être soutenu puissamment par l'État, surtout qu'il répond également à des enjeux écologiques majeurs. Ici même, nous votions, il y a près d'un an, lors de l'examen de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi GEC, un fonds pour le réemploi solidaire, qui a été sérieusement détricoté par le décret d'application et sur lequel les associations du réemploi et nombre de parlementaires de tous bords vous ont alerté. Par ailleurs, ce qu'il reste de ce fonds de réemploi ne sera accessible qu'en 2022. Aujourd'hui, les mêmes parlementaires, unis au-delà des clivages partisans, investis sur ces questions d'économie circulaire, vous invitent à recevoir favorablement notre proposition, qui permettrait de ce secteur indispensable à l'activité, à l'emploi et à la transition écologique. L'adoption de cet amendement permettrait d'assurer la confiance de l'État dans ce secteur, qui est au croisement de multiples enjeux contemporains et répond à la quête de sens recherché par les citoyens : développement de circuits courts, production locale, cohésion sociale. Cet amendement vous donne la possibilité, monsieur le ministre, de reconnaître pleinement le réemploi solidaire comme un secteur stratégique de l'économie française, véritable amortisseur social et environnemental du pays. La parole

un budget de 500 millions d'euros est déjà prévu pour l'économie circulaire et les circuits courts dans le plan de relance. Par ailleurs, l'Ademe dispose de budgets d'intervention

C'est un nouveau cri d'alerte qui était lancé sur la dégradation accrue et extrêmement préoccupante de la situation et des conditions de vie des habitants et du décrochage vis-à-vis de la République dans ces quartiers. Le Président de la République voulait faire des quartiers de la politique de la ville de grands territoires gagnants. Il s'était engagé, dans son discours de Tourcoing, le 16 novembre 2017, à encourager l'ensemble des acteurs et associations qui jouent un rôle fondamental dans les quartiers. Il avait annoncé lui-même la mise en place d'une plateforme mettant en ligne les bonnes initiatives et permettant de les financer, pour les démultiplier dans tous les territoires où elles sont pertinentes. Le groupe socialiste avait d'ailleurs défendu cette position sur ces travées. Qu'en est-il trois ans après ? Nous constatons un manque de confiance à l'égard des élus et acteurs de terrain, un sentiment de non-assistance à territoire en danger. Pourtant, les acteurs locaux font souvent mieux que les pouvoirs publics dans ces territoires, car ils en connaissent la complexité et les fragilités. Il est de la responsabilité de l'État de les soutenir dans leur engagement. Pour accompagner cette mobilisation sans faille des acteurs de terrain, notre amendement vise à créer un conseil national des solutions composé d'élus, d'associatifs, de fonctionnaires, d'entrepreneurs et d'universitaires bénévoles. Il aura vocation à identifier, promouvoir et évaluer les solutions efficaces sur le terrain en matière d'emploi, de citoyenneté, d'éducation, de sécurité, de mobilité et de logement. Il aura également comme première mission de mettre en place des collectifs pour l'emploi et la formation dans les 100 villes les plus pauvres de France. Notre amendement propose 75 millions d'euros pour redonner confiance et espoir aux millions d'habitants qui vivent dans les quartiers les plus en difficulté, 75 millions d'euros pour contribuer à la grande mobilisation nationale annoncée il y a trois ans. Il n'est jamais trop tard ! Le plan de relance doit aussi être l'occasion de redonner vie à la République dans les quartiers de la politique de la ville, pour restaurer la cohésion dans notre pays. Faisons ensemble le pari d'une nouvelle confiance dans nos territoires pour faire gagner la République. Les élus des quartiers demandent le soutien et la confiance du pays. Mes chers collègues, c'est l'appel qui nous est lancé collectivement. Quel est l'avis

Madame Billon, vise à renforcer le soutien aux salles de cinéma, qui sont particulièrement affectées par la crise sanitaire et économique. Une aide exceptionnelle de 100 millions d'euros a déjà été débloquée pour le dernier trimestre de 2020, mais le plan de relance demeure largement sous-dimensionné pour poursuivre ce soutien. Sur les 165 millions d'euros de crédits dévolus dans la mission à la filière cinéma et audiovisuel, seuls 30 millions d'euros devraient en effet revenir aux salles de cinéma. Or leur manque à gagner s'établirait déjà à 1 milliard d'euros. Il vous est ici proposé d'abonder de 70 millions d'euros les aides versées aux salles de cinéma et de porter ainsi leur niveau global à 200 millions d'euros, de façon à pouvoir compenser à hauteur de 20 % les baisses qu'elles subissent. Ce versement complémentaire est indispensable à leur survie économique. Quel

seulement des fortes attentes des citoyens en matière de bien-être animal et d'alimentation de proximité, mais aussi de la nécessaire amélioration des conditions de travail des salariés dans les abattoirs, l'effort financier actuellement prévu par le plan de relance reste largement insuffisant. L'amendement vise ainsi à apporter un soutien aux outils d'abattage adaptés à l'élevage de demain, que ce soit pour les conditions de travail, de relocalisation ou pour la protection animale. Tel qu'il est prévu, le plan de modernisation ne parviendra pas à enrayer la forte diminution en France du nombre d'abattoirs. Les petits abattoirs locaux sont pourtant essentiels pour la relocalisation de l'alimentation, alors que les consommateurs réclament toujours plus de proximité. Le maillage du territoire est également nécessaire pour limiter le transport, ce qui est positif à la fois pour les émissions de CO2 et pour le bien-être des animaux. Il est essentiel que ce plan de modernisation des abattoirs soit dirigé avant tout vers l'amélioration du bien-être animal et des conditions de travail des salariés dans les petits abattoirs de proximité. Cette somme devra également permettre de soutenir l'abattage à la ferme, la mise en place d'abattoirs mobiles, actuellement en expérimentation sur les territoires. Aussi, nous proposons de flécher prioritairement les sommes prévues vers la construction d'un maillage resserré d'abattoir de proximité, respectueux à la fois des animaux et des hommes, et des hommes, en lien avec des filières territorialisées d'élevage durable et en phase avec les attentes sociétales. Monsieur le sénateur Labbé, si la situation économique de nombreux abattoirs locaux est particulièrement tendue, ce qui pourrait justifier un plan de sauvegarde, il faut

Marie-Claude Varaillas. Avec cet amendement, nous voulons revenir sur un sujet qui nous mobilise, à savoir la lutte contre la pratique impitoyable des expulsions locatives. Avant tout, il faut le dire, nous donnons acte à ce gouvernement d'avoir interdit les expulsions locatives durant la période couvrant l'état d'urgence, puis d'avoir donné des instructions aux préfets jusqu'à la reprise de la trêve hivernale, soit au début du deuxième confinement. C'est une bonne chose, même si nous aurions préféré que cette interdiction concerne également l'ensemble de la procédure et, donc, les commandements de payer. L'expulsion n'étant que le bout de la chaîne de l'exclusion, c'est très en amont qu'il convient d'agir. Au regard de la situation sociale particulièrement dégradée, avec des prévisions très sombres en matière de PIB prévisible du nombre de chômeurs, nous considérons qu'il convient de proroger cette suspension des expulsions locatives, alors que nos concitoyens vont se trouver en grande fragilité, les chiffres le rappellent, et que les associations sont particulièrement inquiètes. Les plus fragiles sont les grands oubliés de ce plan de relance, alors même que la pandémie a renforcé les inégalités et précipité dans la pauvreté dans la pauvreté trop de nos concitoyens. Selon les spécialistes, l'année 2020, pandémie oblige, devrait faire exploser le taux de pauvreté. Le volume des demandes d'allocation de RSA, nous l'avons vu, bat tous les records et dépasse les 3 000 par jour. par jour. Selon le Secours catholique, l'année 2020 est l'année de tous les dangers pour ces publics. Évidemment, nous ne pouvons nous y résoudre. Déjà, en 2019, les expulsions locatives avaient battu tous les records, avec pas moins de 16 700 Le chiffre de 2021 sera terrible sans engagement fort de la Nation tout entière. Je vous rappelle cet autre chiffre que nous a donné récemment la Fondation Abbé Pierre : 300 000 personnes se trouvent déjà sans domicile personnel. Pour cette raison, nous vous demandons, avec les associations luttant contre le mal-logement, le maintien de la trêve hivernale jusqu'au 31 octobre 2021, en confirmant les instructions données aux préfets dans la période précédente de ne pas pratiquer d'expulsions locatives sans relogement.

En effet, le Président de la République a déclaré qu'il souhaitait atteindre 30 % de territoires naturels d'ici à la fin de son mandat. On en est encore loin ! Si l'on souhaite atteindre 10 % d'espaces sous protection d'ici à 2022, il va falloir y mettre d'autres moyens, à la fois financiers et humains.

Il y a une vraie attente sur la conservation de la biodiversité. Cet abondement par un montant alloué aux aires protégées irait vers les parcs naturels parcs naturels régionaux, les parcs naturels marins et les conservatoires, ce qui permettrait d'avoir une vraie politique en matière d'acquisitions foncières, de restauration, de gestion des écosystèmes

l'avis de la commission ? Monsieur Gontard, les crédits du plan de relance s'ajoutent aux crédits prévus par le programme 113 pour accélérer les actions mises en oeuvre dans ce cadre.

tout en fléchant ces moyens vers les filières de qualité, dont l'agriculture biologique. Actuellement, le plan de relance ne prévoit que peu de garanties environnementales sur les filières qui seront soutenues par le plan Protéines. La hausse du budget proposée par La hausse du budget proposée par cet amendement vise à soutenir les filières de qualité- AOC, IGP -et biologiques. Il s'agit notamment de soutenir les légumes secs à destination de l'alimentation humaine, qui ont un clair avantage concurrentiel par rapport aux filières conventionnelles concurrencées par les importations. On connaît notre dépendance aux protéines végétales importées en masse d'Amérique du Sud. Le ministre de l'agriculture a annoncé la mise en oeuvre du plan Protéines national, qui a été pensé depuis 2009. Enfin, on y arrive ! La demande est forte actuellement pour des élevages qui consomment des protéines végétales bio,

Dantec. Cet amendement vise à abonder le volet forêt du plan de relance de 50 millions d'euros. Nous le savons tous, la forêt a besoin d'investissements publics forts pour soutenir une sylviculture adaptée aux enjeux climatiques et sociétaux, pour restaurer la biodiversité du territoire

les montants actuellement prévus par le texte sont insuffisants. Le présent amendement vise également à appeler l'attention sur les nécessaires conditionnalités à apporter au plan Forêt. C'est un point sur lequel je veux insister. En effet, des pratiques de monoculture ou des coupes rases massives ne doivent plus être soutenues. Elles sont souvent inadaptées aux enjeux climatiques et font l'objet de contestations sociales. À cet égard, il faut noter que la Convention citoyenne pour le climat a proposé dans son rapport l'encadrement des coupes rases. Des pratiques de diversification, de recherche et d'expérimentation sur l'évolution de la forêt, des itinéraires techniques alternatifs, le renouvellement par régénération naturelle doivent être soutenus pour permettre le développement d'une forêt résiliente, espace de biodiversité et de production durable. En tant que président

est à M. Joël Labbé. Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d'euros le budget consacré à la préservation et à la reconquête des haies. Il est en effet nécessaire de renforcer ce budget pour faire face aux enjeux de la transition agroécologique en accompagnant les agriculteurs. Les haies ont un impact agronomique et environnemental majeur non seulement d'améliorer la qualité du sol et de limiter l'utilisation d'engrais, mais aussi de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, notamment en abritant les auxiliaires de culture. Leur rôle pour la préservation de l'eau et des sols n'est donc plus à démontrer. Elles ont aussi un impact pour le climat, notamment en favorisant le captage de carbone dans le sol. De plus, les haies constituent un gisement important d'énergies renouvelables. Elles ont enfin un fort intérêt pour les paysages et pour la biodiversité.

qui disparaissaient chaque année, malgré la réglementation, d'où la nécessité d'inciter véritablement à la préservation des haies existantes et à l'implantation de nouvelles.

d'implanter 7 000 kilomètres de haies, ce qui est une belle performance quand on part de zéro. C'est à peu près 70 kilomètres par département. Vous l'avez dit à juste titre, il faudrait déjà éviter de détruire les haies

vise à augmenter de 50 millions d'euros le montant prévu pour les projets alimentaires territoriaux dans le plan de relance. le plan de relance. En effet, ce sont des outils efficaces de relocalisation de l'alimentation sur les territoires, aujourd'hui encore trop peu développés, notamment à cause d'un manque de financement. Les attentes sociétales en matière de qualité et de relocalisation de l'alimentation, la nécessité de prix agricoles justes pour les producteurs et éleveurs et la prise en compte des enjeux environnementaux appelleraient pourtant leur généralisation. Avec cet amendement, nous proposons donc d'abonder de 50 millions d'euros les crédits dédiés aux collectivités territoriales pour accélérer la transition agroécologique de l'action n° la commission ?

pour explication de vote. Il y a quand même urgence. N'oublions pas que nous avons voté, pour la restauration collective, une obligation à 50 % de produits locaux de qualité,

d'activité partielle en Nouvelle-Calédonie. L'économie calédonienne a elle aussi été fortement touchée par les mesures consécutives à la crise sanitaire. Pour endiguer la spirale de la pauvreté, le Gouvernement calédonien a donc, comme en métropole, déployé un dispositif de chômage partiel.

En effet, cet emprunt va entraîner un alourdissement de la fiscalité locale à peine soutenable pour les Calédoniens, dans une phase où les efforts financiers devraient plutôt être fléchés en faveur des investissements nécessaires à la relance économique. À l'heure où l'Union européenne finance substantiellement la politique du chômage partiel en France, alors qu'elle n'en a pas formellement la compétence, il semble souhaitable que l'État transcende le strict cadre de la répartition de la compétence en matière économique pour financer le dispositif d'accès Je suis défavorable à cet amendement, qui vise à mobiliser près de 42 millions d'euros en faveur de la Nouvelle-Calédonie, spécifiquement affectés au financement du chômage partiel dans ce territoire. Les salariés en Nouvelle-Calédonie ne bénéficient pas du chômage partiel national. S'agissant d'une prestation relevant d'une logique assurantielle, il est impossible de l'étendre à la Nouvelle-Calédonie. Cet amendement est donc, selon moi, inopérant. La Nouvelle-Calédonie a d'ailleurs mis en oeuvre, à compter de mars, une allocation covid pour pallier cette difficulté. Il convient de relever que ce problème concerne la Polynésie française également. Enfin, le soutien de l'État à la politique menée par la Nouvelle-Calédonie repose d'ores et déjà

est de 1 600 euros en moyenne, cette somme permettant de financer l'accompagnement mis en place. À l'occasion du présent plan de relance, davantage de

Face à cette situation, nous n'avons pas forcément les mêmes réponses. Moi, je suis convaincue que la garantie jeunes est un bon dispositif, pas seulement parce qu'il offre une allocation pour l'ensemble des jeunes-

que le Gouvernement reconnaît comme une bonne solution, puisqu'il a préconisé l'augmentation de 100 000 à 150 000, et bientôt à 200 000, de leur nombre. Néanmoins, il y a un vrai sujet sur les fonds attribués aux missions locales pour la mise en oeuvre de cet accompagnement, qui est la clé de la réussite de la garantie jeunes et, donc, du Pacea. Comme l'a justement dit notre collègue collègue Raynal, il y a une différence entre les financements de base, dans le cadre du programme 103, à hauteur de 1 600 euros par jeune, et ceux octroyés dans le cadre du plan de relance, l'aide donnée aux missions locales n'étant que de 940 euros par jeune, ce qui risque d'entraîner un accompagnement dégradé.

de favoriser le développement d'activités de montagne respectueuses de l'environnement. Ainsi, nous proposons de dédier un fonds de 15 millions d'euros par an, sur une période de deux ans, aux stations de ski qui n'ont pas pu ouvrir plus de cent jours lors de chacune des cinq dernières saisons d'hiver.

à la demande du groupe socialiste, a créé une commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols

savoir la création d'un fonds national spécifiquement dédié à la sécurisation et à la réhabilitation des sites orphelins industriels et miniers, placé sous la gestion de l'Ademe.

de cet amendement, nous entendons remédier aux difficultés de financement de la réhabilitation des sites pollués, puisque les collectivités ne peuvent pas faire face à cette tâche.

Le combat pour les biens communs doit être au coeur de cette relance. L'eau est une ressource qui se raréfie, qui fait souvent l'objet de conflits politiques, ou géopolitiques, et dont la gestion est en France encore largement confiée au Les régies publiques permettent un meilleur service, un contrôle démocratique de la ressource et, souvent, une baisse de prix ou une tarification sociale, du fait de la suppression de la marge prise par les multinationales. Cependant, les collectivités françaises rencontrent souvent l'opposition ferme des entreprises qui contrôlent actuellement la ressource. pendant des décennies d'une rente confortable et font tout pour la conserver. Les collectivités sont parfois menacées de devoir mener des travaux importants et d'engager des investissements d'ampleur pour reprendre ou reconstruire les réseaux appropriés. Cet amendement vise donc à créer un dispositif de soutien aux collectivités qui s'engagent dans la création d'une régie publique de l'eau. L'accès à une eau de qualité contrôlée démocratiquement sera l'un des combats importants des années à venir. C'est pourquoi les écologistes proposent également de rendre l'eau

soit parce que le système des syndicats intercommunaux rend presque impossible la sortie de ces syndicats. J'en veux pour preuve les nombreuses collectivités de l'Île-de-France, notamment dans les départements du Val-de-Marne et de l'Essonne,

! Nous nous privons là du libre choix des collectivités locales et nous les empêchons d'investir aussi massivement qu'elles le souhaitent, pour une politique de l'eau plus conforme à l'environnement et à l'intérêt public.

ou les intercommunalités sont en mauvais état. Ces 20 millions d'euros ne seront donc vraiment pas de trop pour améliorer la situation.

de 10 millions d'euros en crédits de paiement, dédiée au soutien du déploiement d'applications industrielles de la 5G en France. La modernisation de l'industrie française doit figurer parmi les axes prioritaires de la relance. En effet, l'outil industriel français est en moyenne deux fois plus ancien que son équivalent allemand bien moins robotisé et bien moins digitalisé. Les années 2020 et 2021 sont deux années charnières pour le déploiement de la 5G en France. L'arrivée de la 5G et des technologies liées- liées- objets connectés, monitoring, réalité augmentée -risque de creuser encore l'écart de compétitivité entre les entreprises industrielles françaises et leurs concurrentes si un effort particulier n'est pas consenti pour soutenir le déploiement de la 5G dans les usines et son intégration au sein des processus de production. Cet amendement vise donc à ouvrir une ligne de financement supplémentaire et spécifique qui permettrait la mise en place d'un guichet de subvention par lequel l'État cofinancerait le déploiement de solutions industrielles utilisant la 5G, notamment dans les TPE et PME industrielles, dans une optique de modernisation rapide de l'industrie française.

est l'avis du Gouvernement ? Défavorable. Monsieur Montaugé,

Cet amendement, le troisième que je présente pour soutenir les initiatives culturelles, vise à amorcer des changements structurels du secteur et des territoires vers un modèle plus solidaire, plus durable et plus respectueux des droits humains. La crise que nous traversons est un défi pour le monde de la culture. Elle en menace les acteurs, mais peut aussi être l'occasion de se réinventer et d'engager une réelle transition : tel est le sens de la relance culturelle que nous voulons impulser. Nous proposons donc de créer un fonds pour la transition urbaine et rurale, doté de 20 millions d'euros par an. Ce programme s'appuie sur une convention d'objectifs et de moyens qui décline des actions sur deux ans, autour de trois axes : renforcer les coopérations, développer la solidarité financière et soutenir l'expérimentation. Nous voulons le faire de manière transversale ; ce programme pourra s'appuyer sur des partenariats actifs et financiers avec des acteurs du financement solidaire de l'accompagnement, de la formation et de la recherche. On se plaît à rappeler que le Sénat est la chambre des territoires. Il est temps de le prouver aujourd'hui en soutenant cette initiative, qui permettra d'ancrer localement les projets culturels dans une logique d'écosystème, afin de redynamiser toute une économie locale de la culture, qui, par essence, est non délocalisable.

Le soutien aux industries culturelles et au maillage culturel des territoires fait l'objet d'une dotation quasiment équivalente à celle qui est proposée par le présent amendement. Ainsi, 14 millions d'euros sont prévus en faveur de l'Ifcic, afin de soutenir des projets innovants. Par ailleurs, la mise en place de quartiers culturels et créatifs, en particulier dans des centres urbains dévitalisés, serait dotée de 3 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 1,5 million d'euros

à très faible impact en gaz à effet de serre et à impact positif pour la biodiversité. Dans leur proposition, les citoyens ont ainsi demandé la restauration de l'aide au maintien en agriculture biologique, ce que nous-mêmes réclamons depuis longtemps. depuis longtemps. En effet, en septembre 2017, le Gouvernement a annoncé l'arrêt du financement par l'État de l'aide au maintien en agriculture biologique. Trois ans plus tard, là où les régions n'ont pas pris le relais- il en les agriculteurs bio n'ont plus accès à cette aide, ce qui pénalise le développement de la filière. Pourtant, la demande de produits biologiques continue d'augmenter, et le dernier rapport de France Stratégie sur les performances économiques et environnementales de l'agroécologie affirme, une fois encore, l'efficacité de l'agriculture biologique, définie comme « la plus performante d'un point de vue économique et environnemental aujourd'hui ». Cet amendement vise donc à affecter 20 millions d'euros à un nouveau programme « Aide au maintien en agriculture biologique », destiné à rétablir le financement par l'État de l'aide au maintien. Je voudrais vous rappeler, monsieur

Le revenu de base peut répondre à cette problématique dans un contexte de précarisation des trajectoires d'emploi, renforcée par la crise économique actuelle. Le présent amendement vise à budgéter une expérimentation de ce dispositif pour l'ensemble des conseils départementaux qui le souhaiteraient, pour un coût total de 18 millions d'euros.

relance, un fonds d'aide de 10 millions d'euros dédié à la modernisation et à la diversification des stations-service réparties sur le territoire national. Parmi les 11 068 stations-service situées en France,

leurs investissements, pourtant essentiels à la survie des entreprises, à la continuité de l'activité de distribution de carburants, ainsi qu'à l'investissement dans les énergies propres et à la mise aux normes environnementales. Cet amendement vise à ajouter 10 millions d'euros au programme « Écologie » de la mission « Plan de relance », à l'action n° 07, Infrastructures et mobilités vertes. Pour ce faire, un retrait de 10 millions d'euros est effectué dans le programme n° 363, « Compétitivité à l'action n° 02, Souveraineté technologique et résilience. Cette répartition permet de favoriser le soutien aux stations-service, tout en pénalisant le moins possible les objectifs de compétitivité

pour contribuer activement au développement des filières protéines végétales des actions menées au plus près des besoins des agriculteurs et des consommateurs. Les Civam, les GAB, les Adear, les Cuma,

Il est essentiel de leur permettre de participer à une transition protéique prenant en compte les enjeux sociaux, agronomiques, environnementaux et économiques des territoires. Quel est l'avis de la commission

Les 680 radios de territoires en France métropolitaine et outre-mer, à statut associatif, ont poursuivi leurs programmes au bénéfice des populations et des services de l'État dans des conditions budgétaires dramatiques. Elles ont été unanimement saluées, depuis le premier jour du confinement et jusqu'à présent. La perte moyenne est à ce stade estimée à 27 000 euros par radio locale, à laquelle il faut ajouter l'impact systémique sur les barèmes des subventions réglementaires en 2021 et 2022. l'organisation professionnelle majoritaire des radios associatives indique une perte d'emplois pouvant aller jusqu'à un équivalent temps plein par entreprise, soit près de 700 emplois Cette catégorie de radios, avec ses deux millions d'auditrices et d'auditeurs, constitue un secteur professionnel spécifique de l'audiovisuel relevant de l'économie sociale et solidaire. Ce secteur est fort de 680 très petites entreprises, associations loi 1901, et de 2 600 salariés, dont 300 journalistes. loi de finances rectificative a accordé une aide spéciale de 30 millions d'euros aux radios et télévisions, quelle que soit la nature de leur programmation et indistinctement de leur statut, commercial ou non.

Afin de rendre l'amendement recevable, il est proposé de compenser les crédits alloués par une annulation d'un montant équivalent de crédits à l'action n° 04 du programme n°

un mécanisme de collecte de l'épargne et de financement des investissements cloisonnés, qui échapperait au court-termisme dévastateur des marchés financiers et soutiendrait la transition écologique.

et en accord avec la commission des finances, je vous propose de reporter l'examen des articles rattachés aux missions « Plan de relance » et « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » à samedi prochain. Ce report entraînera une réorganisation de l'ordre d'examen des missions de l'après-midi et du soir, en concertation avec la commission des finances et le Gouvernement. Afin de pouvoir disposer du temps nécessaire pour cette réorganisation, l'ordre du jour définitif sera fixé demain matin. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. Voici quel sera